Monsieur le président,

des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 vient juste de s'achever, est parvenue à un accord. Afin de permettre le dépôt et la diffusion du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je vais toutefois devoir suspendre la séance.

Monsieur le président,

La séance est reprise. Monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est avec une profonde émotion que nous avons appris le décès hier de notre ancien collègue Jacques Oudin, qui fut sénateur de la Vendée de 1986 à 2004. Conseiller général du canton de Noirmoutier-en-l'Île, vice-président du conseil général de la Vendée, conseiller municipal de La Guérinière, Jacques Oudin fut l'un des piliers de la vie politique vendéenne. Il participa activement au développement de son département, et notamment de l'île de Noirmoutier, grâce à ses nombreuses contributions au sein de l'association vendéenne des élus du littoral. Élu sénateur de la Vendée en 1986, Jacques Oudin appartenait au groupe du Rassemblement pour la République. J'eus le plaisir de partager avec lui nombre de réunions de notre groupe et de journées parlementaires. Pendant ses deux mandats, il fut un membre éminent de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, dont il fut secrétaire, puis vice-président. La commission bénéficia des compétences de ce magistrat de la Cour des comptes et de cet ancien membre du cabinet d'Olivier Guichard, ministre de l'aménagement du territoire. Président fondateur du Cercle français de l'eau, Oudin s'engagea en faveur de la coopération décentralisée dans le domaine de l'eau. Il créa, en tant que sénateur, le groupe d'études et participa à l'élaboration de la troisième loi sur l'eau. Sa mère, qui lui donna la vie sur un bateau, quelque part en mer de Chine, marqua profondément l'existence de ce gaulliste vendéen. Son engagement au sein du groupe d'amitié France-Vietnam n'en fut que plus grand. J'avais, comme un certain nombre d'entre nous, noué avec Jacques Oudin, pendant ses mandats et au-delà, de solides liens d'amitié. Nous appréciions son intelligence et sa gentillesse. Je le revois encore, attentif et passionné, assister aux réunions et aux colloques organisés par l'amicale gaulliste du Sénat, dont il fut secrétaire général, et prendre, encore et toujours, des photos- c'était sa spécialité. Je le revois lors de nos moments de ressourcement à Colombey-les-Deux-Églises, autour de la figure de notre histoire qui donna sens à son engagement : le général de Gaulle.

Au nom du Sénat, je souhaite exprimer notre sympathie et notre compassion à son épouse, Anne-Marie, à qui j'ai parlé au téléphone, à sa famille, à ses proches, à ses compagnons, ainsi qu'au président- Vendéen, lui aussi -et aux membres du groupe Les Républicains. Je vous propose d'observer un moment de recueillement.

jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19

En ce moment difficile pour la Nation, le Parlement joue pleinement son rôle, qui est de concilier le respect des principes démocratiques et la prise en compte de l'urgence sanitaire. L'un ne peut aller sans l'autre.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les travaux de la commission mixte paritaire, qui se sont engagés ce matin et se sont prolongés jusqu'à ont été particulièrement riches et intenses. Chacun des membres de la commission mixte paritaire était pleinement imprégné de la responsabilité qui nous incombe collectivement : parvenir à un accord, sans compromettre les convictions que nous avons à défendre, mais avec l'idée que l'intérêt général commande de manifester l'union de la représentation nationale aux côtés du Gouvernement. Naturellement,

la nécessité de donner au Gouvernement les moyens d'action dont il a besoin pour combattre le fléau qui accable notre pays, comme beaucoup d'autres, depuis plusieurs semaines.

Nous voulions également éviter de prendre des mesures dérogatoires au droit commun dépassant les exigences du combat contre le Covid-19.

Nous nous sommes concentrés sur la lutte contre le Covid-19, et nous n'avons pas voulu préjuger des moyens qui seraient nécessaires si d'autres fléaux sanitaires accablaient notre pays dans plusieurs années. Le régime de l'état d'urgence sanitaire est donc temporaire.

Les pouvoirs donnés au Gouvernement sont importants, parce qu'il faut pouvoir limiter la liberté d'aller et venir. Il faut pouvoir limiter la liberté de réunion. Il faut pouvoir aussi limiter la liberté d'entreprendre. Mais- vous vous en souvenez, puisque l'état d'urgence est dans tous les esprits, pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme -, la loi de 1955, qui permet, pour des motifs de sécurité, de déclarer l'état d'urgence, énumère les catégories de mesures susceptibles d'être prises périmètre de sécurité, perquisitions administratives, assignation à résidence, fermeture de lieux de culte salafiste, etc. Toutes ces

faire en sorte que le Gouvernement dispose de pouvoirs importants, mais éviter qu'il ne porte trop fortement atteinte à nos libertés. J'y insiste : des atteintes aux libertés sont nécessaires, mais elles doivent être strictement limitées. Nous avons donc exclu que le Gouvernement puisse prendre des mesures d'ordre général en dehors de la liste que nous avons fixée, quand elles portent atteinte à la liberté d'aller et venir et à la liberté de réunion. En revanche, nous avons accepté qu'il puisse prendre des mesures, dont nous n'avons pas défini exactement les contours, qui seraient susceptibles de porter atteinte à la liberté d'entreprendre. Ces mesures, on peut les imaginer en prenant comme référence l'organisation de la Nation en temps de guerre,

Il faut que le Gouvernement puisse produire des masques, il faut qu'il puisse produire des respirateurs artificiels, il faut qu'il puisse produire les équipements, les matériels, les médicaments et, éventuellement, qui seront nécessaires à l'efficacité de la lutte contre cette épidémie. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté de lui laisser la prérogative de prendre ces mesures. Toutefois, il ne pourra le faire que par décret du Premier ministre, et non par simple arrêté du ministre de la santé, et ce décret pourra être déféré au Conseil d'État, lequel devra se prononcer

du report du second tour de l'élection municipale dans plus de 5 000 communes de France. Nous ne pouvions pas ne pas les traiter. Ce n'est pas nous qui les avons inscrites à l'ordre du jour : c'est la situation née du report du second tour des élections municipales qui nous imposait d'en parler.

-que les maires de France sachent comment s'y prendre, n'aient pas de doute quant au fait qu'ils ont la pleine responsabilité de leur commune pour mener à bien leur mission de maire. Ce n'est pas facile de concevoir ce qui n'a jamais été fait, en l'occurrence comment organiser le travail des communes quand, dans celles-ci, le second tour n'a pas eu lieu. Nous avons prévu des règles simples : quand le second tour n'a pas eu lieu, les anciens maires et les anciennes équipes continuent à agir. La règle est claire. Tous les Français doivent la connaître. Ces élus vont continuer à agir jusqu'à ce que nous puissions mettre en place les nouvelles équipes. Comme, par ailleurs, nous n'avons pas réussi à élire les maires, ce dimanche, hier et avant-hier,

l'élection est définitive, elle ne pourra jamais être remise en cause. C'est écrit dans ce texte. Les équipes n'ont pas pu se mettre en place ce week-end, mais c'est seulement leur entrée en fonctions

des mesures permettant d'élire les maires, parce que c'est très important pour la République, en recourant au vote par correspondance, au vote à l'urne, voire au vote électronique. Comme nous ne pouvons pas improviser les modalités d'organisation de ces formes d'expression du vote, nous demandons au Gouvernement de prendre ces mesures dans les semaines qui viennent. Je le répète, même si le confinement continue, on pourra élire les maires.

possible, afin de pouvoir tenir compte de l'évolution de la situation sanitaire. Nous avons donc décidé qu'un rapport du comité scientifique sera publié

on ne pourra plus geler le premier tour : on ne saurait préjuger que les électeurs du premier tour du mois de mars n'ont pas changé d'avis six mois plus tard ! Ce serait restreindre leur liberté de vote ; ce serait contraindre le suffrage universel. Nous écrivons noir sur blanc

monsieur le président de la commission mixte paritaire, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis ce dimanche pour l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est tenue tout à l'heure. Avant toute chose, je tiens à saluer, monsieur le président, la mobilisation exceptionnelle du Sénat, de ses élus, de ses fonctionnaires et collaborateurs, pour que la continuité de nos institutions soit assurée et que le débat démocratique existe en ces temps difficiles. Vous me permettrez aussi de remercier les services du Gouvernement qui ont contribué à l'écriture de ce projet de loi et des ordonnances à venir. Ce débat, qui nous a tous pleinement mobilisés, a eu lieu alors même que des règles sanitaires très strictes été édictées au sein même de votre assemblée. Nous nous y sommes collectivement pliés avec discipline, de la même manière que nos concitoyens appliquent au quotidien les consignes sanitaires du Gouvernement. Il en allait, vous l'avez dit, monsieur le président, de notre devoir d'exemplarité. Je souhaite également souligner la qualité du dialogue entre les deux assemblées et le Gouvernement pour parvenir à examiner dans des conditions satisfaisantes pas moins de trois projets de loi entre jeudi et aujourd'hui. Aucun examen rapide ne peut être sérieux s'il n'existe pas un consensus de toutes les parties prenantes sur l'urgence d'agir et sur les réponses à apporter. Il est indéniable qu'il y a eu entre nous et vous des divergences. Certaines demeurent, et c'est normal. Cela prouve que notre démocratie n'est pas mise entre parenthèses. Nous les avons surmontées, c'est la fonction du débat parlementaire. Je voudrais, à ce titre, vous remercier, monsieur le président, pour votre disponibilité, votre écoute et votre rôle essentiel dans la conciliation des différentes parties prenantes pour créer les conditions d'un débat démocratique nécessaire et favoriser les consensus. Je salue également l'engagement du président de la commission des lois ainsi que celui des présidents de groupe de votre assemblée, qui ont toujours accepté de dialoguer et d'avancer quels que soient les obstacles, avec un très grand esprit de responsabilité. Nombre de citoyens pourraient s'étonner que le Parlement ait eu besoin de quatre jours pour adopter une loi dite « d'urgence » destinée à faire face à l'épidémie de Covid-19, alors qu'ils sont eux-mêmes confinés chez eux et que, hélas, ils sont inquiets pour leurs proches, quand certains ne sont pas endeuillés. Nous devons assumer ce débat que nous avons tous voulu et appelé de nos voeux, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous restons convaincus que le débat parlementaire éclaire toujours l'opinion publique et que les Français attendent une réponse claire et forte sur ce que l'État va faire dans les prochaines semaines. La deuxième, c'est que ce débat était une oeuvre utile de transparence sur la situation économique, sanitaire et sociale. La troisième, enfin, c'est que le consensus autour de mesures exceptionnelles rend d'autant plus fortes sa compréhension et son acceptation par nos concitoyens. Nos débats ont montré tout l'intérêt de la démocratie représentative vous avez fait remonter les observations, les interrogations, les inquiétudes de nos concitoyens sur le terrain, et nous avons voulu y apporter des réponses. Je n'oublie pas le rôle essentiel de vos collègues, absents de l'hémicycle en raison des règles strictes qui ont été édictées et que nous nous sommes imposées, mais dont vous avez relayé, je le sais, les attentes. Je voudrais, par votre intermédiaire, les remercier et saluer leur engagement exceptionnel dans leurs territoires. Ils jouent pleinement leur rôle, chaque jour, auprès de leurs concitoyens. Plus précisément, je voudrais, à la suite du président de la je voudrais, à la suite du président de la commission mixte paritaire, revenir sur quelques mesures de ce texte. Le titre II sur l'état d'urgence sanitaire donne les moyens au Gouvernement et à ses représentants de prendre des mesures réglementaires fortes pour enrayer la propagation du Covid-19, en s'inspirant notamment de la loi du 3 avril 1955. Les mesures exceptionnelles qui pourront être prises ne se feront évidemment pas sans contrôle si les circonstances exigeaient qu'elles soient mises en oeuvre. Le Parlement devra autoriser par la loi la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, la décision d'y recourir devra être éclairée par des données scientifiques rendues publiques. Tant l'Assemblée nationale que le Sénat pourront requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. S'appuyer sur la science pour prendre nos propres responsabilités politiques et poursuivre le contrôle de l'action du Gouvernement dans cette période exceptionnelle sont des choses précieuses. Outre des mesures plus coercitives à l'encontre de multirécidivistes contribuant à la propagation du virus par leur comportement irresponsable, des décisions de bon sens ont été prises dans le débat entre l'Assemblée nationale Le titre III nous dote collectivement d'un arsenal à même de répondre notamment à la situation économique détériorée par la crise sanitaire. Environ quarante habilitations sont prévues. C'est un choix radical que le Gouvernement assume. Il faut être humble : nous ne connaissons pas aujourd'hui toutes les mesures qui seront à prendre en fonction de l'évolution de la situation. Mais, d'ores et déjà, nous prévoyons le soutien massif à la trésorerie des entreprises et des aides directes ou indirectes à ces dernières. Le droit du travail sera aussi temporairement adapté afin de garantir de la souplesse pour limiter les ruptures définitives de contrat de travail. Ces mesures temporaires auront pour seul et unique objectif de permettre la poursuite du travail pour subvenir aux besoins essentiels de la Nation. D'autres dispositions, qui pourront être complétées par ordonnance, sont de nature à adapter les procédures du quotidien, auxquelles nous ne prêtons pas toujours attention en période normale : je pense au fonctionnement des organes des collectivités territoriales, à celui des syndics de copropriété, aux procédures judiciaires. C'est là aussi que le débat parlementaire a pris tout son sens rappeler au Gouvernement tel pan de notre vie en collectivité qui mérite que soit prise une mesure en particulier ou une autre. Enfin, le titre III tire les conséquences de la décision du report du second tour des élections municipales et prévoit les modalités d'installation des conseils municipaux élus au premier tour. Je ne reviendrai pas sur ces dispositions, le président de la commission mixte paritaire les ayant très bien explicitées, si ce n'est pour me féliciter qu'un accord ait pu être obtenu entre les deux assemblées sur la question du dépôt des listes en particulier. Ce ne pouvait être, dans cette situation de crise et devant les Français, un point bloquant pour obtenir cet accord conclusif. Ce projet de loi nous donne d'importants moyens pour répondre aux problèmes posés par la propagation du Covid-19. Il ne résoudra pas tout, et il sera sans doute amené à être complété par d'autres dispositions. Nous pouvons nous féliciter du travail accompli ces quatre derniers jours, mais la crise que nous connaissons nous oblige à l'humilité. Cela fait partie de la transparence et, au fond, de la responsabilité. Vous me permettrez de conclure en vous disant, ce que, je crois, nous partageons tous, qu'il faut saluer celles et ceux qui aujourd'hui soignent nos concitoyens, avec professionnalisme et dévouement comme ils l'ont toujours fait, mais plus encore aujourd'hui, celles et ceux qui assurent chaque jour encore la continuité de la vie économique essentielle, la continuité de l'État et la continuité des services dans les collectivités territoriales. À cet égard, vous me permettrez de saluer l'ensemble des élus locaux, qui sont aussi pleinement mobilisés, de saluer l'engagement sans faille des policiers, gendarmes et pompiers, qui veillent à ce que les mesures sanitaires soient scrupuleusement respectées, et des maires aux côtés de nos concitoyens en ces circonstances particulières. Je salue tous ceux qui, par les plus modestes des gestes, constituent un chaînon admirable. Il nous faut plus que jamais leur rendre hommage : nous leur devons déjà beaucoup et nous leur devrons beaucoup. Ils prennent leur part, grande, lourde

Avant de donner la parole à ceux de nos collègues qui sont inscrits dans la discussion générale, je voudrais saluer et remercier le rapporteur de la commission mixte paritaire, René-Paul Savary, qui a oeuvré conjointement avec le président Philippe Bas et ses autres collègues à cette conclusion positive de notre commission mixte paritaire. Merci, monsieur le rapporteur

Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes loin d'être au bout du chemin. Plus que jamais, nous devons affirmer notre solidarité totale à l'égard des soignants et de toutes celles et de tous ceux qui se donnent tellement de mal pour lutter partout contre ce fléau. Nous

dès lors que sont mises en oeuvre les mesures les plus efficaces possible pour lutter contre ce fléau. Nous savons que ces mesures sont nécessairement exceptionnelles.

des initiatives, du comportement et du dévouement de chacun et de chacune d'entre nous. Mes chers collègues, M. le président Philippe Bas vient d'évoquer notre commission mixte paritaire, qui s'est déroulée dans un climat serein.

dans le même temps, notre groupe tient à réaffirmer, en tout point et en toutes circonstances, même exceptionnelles, son attachement aux libertés, son attachement aux droits du Parlement, qui sont constitutifs de l'esprit républicain et de la République. La parole

les familles endeuillées, les personnes malades, les entourages inquiets. J'ai une pensée particulière aussi pour nos collègues sénateurs et tous les collaborateurs du Sénat qui sont ou ont été infectés par le virus. cela fait maintenant trois jours- oui, trois jours ! -que le Parlement débat de ce projet de loi dit « d'urgence ». C'est l'honneur de notre démocratie que de préserver les principes de notre État de droit dans toutes les circonstances, même les plus exceptionnelles, les plus tragiques, les plus éprouvantes pour notre pays. Tout comme Clemenceau avait toujours tenu à ce que le Parlement siégeât durant son ministère, pendant la Grande Guerre. Mais, devant l'urgence sanitaire, économique, sociale et sécuritaire absolue, il s'agissait de ne pas ressembler aux Byzantins, qui dissertaient sur le sexe des anges alors que les Ottomans assiégeaient leur cité. Les débats se sont donc étirés au moment où nos personnels soignants effectuent un travail exceptionnel, dans des conditions épouvantables, eux qui méritent bien plus qu'une série d'hommages, même justifiés. Trois jours de débat, c'est sûrement beaucoup pour nos concitoyens, qui, pour la plupart, ont maintenant pris la mesure de la gravité de la situation. Trois jours pour discuter de points de droit qui peuvent paraître finalement secondaires aux yeux de nos concitoyens au regard des urgences du moment. Monsieur le ministre, nul ici ne doute de l'engagement collectif du Gouvernement. Nous savons que le ministre de la santé mobilise tous les moyens pour que notre système de santé soit en mesure d'absorber le pic épidémique attendu dans quelques jours. Les leçons à tirer seront pour plus tard. L'heure n'est pas à la politique partisane, mais bien à l'unité nationale, et vous pouvez compter évidemment sur le groupe du RDSE dans ce moment. Chacun détient une part de la responsabilité collective qui permettra de lutter efficacement contre l'épidémie. Il y a, bien sûr, les inconscients, qui confondent confinement et vacances. Ceux aussi qui sont allés rejoindre leur résidence secondaire au risque d'étendre la contamination. Mais je voudrais surtout retenir les initiatives remarquables de beaucoup de nos concitoyens, remettant du lien social et de la solidarité au coeur de la cité ici, un supermarché qui réserve des créneaux horaires aux personnes âgées ; là, un maire qui demande à ses administrés de se mobiliser pour rompre l'isolement des résidents d'un Ehpad en leur envoyant des messages ; un autre qui renforce le portage des repas ; un peu partout, une attention à distance retrouvée envers sa famille, son cercle amical ou son voisinage, pour égayer le confinement ou s'assurer que tout va bien. À cet égard, nous souscrivons bien sûr à la création et à la mise en oeuvre immédiate de l'état d'urgence sanitaire. Il y a encore trop de nos compatriotes qui n'ont pas conscience de ce que nous vivons. La pédagogie doit vite le céder à la coercition, au nom de l'intérêt général

En effet, de fortes interrogations demeuraient dans le domaine du droit du travail, où les circonstances exceptionnelles ne peuvent en aucun cas être le prétexte à une régression. Oui, nos deux assemblées ont longuement débattu des modalités de report du second tour des élections

lorsqu'ils savent qu'ils ne seront plus en place dans quelques semaines, mettant en place des mesures importantes comme des plateformes de soins ou des chaînes de solidarité. Partout, avec les agents des collectivités territoriales, ils assurent la continuité des services publics essentiels à la population avec la meilleure qualité possible.

Les ordonnances sont le meilleur moyen de décliner rapidement ces aides secteur par secteur. Mes chers collègues, une fois passé l'état de sidération dans lequel notre pays, à l'instar du monde entier, est plongé, il sera temps de s'interroger et d'analyser ce qui aurait pu être fait autrement. Il faudra aussi, bien sûr, tirer des leçons profondes pour notre système de santé, nos industries stratégiques, notre modèle économique ou encore notre résilience alimentaire. Le groupe du RDSE avait d'ailleurs présenté des propositions fortes à ce sujet.

répondre en droit et dans des délais réduits, pour assurer la continuité de la vie nationale, à une urgence imposée par de tristes circonstances de fait. Plusieurs écueils étaient face à nous confondre réactivité et précipitation et être pris de « démangeaisons législatives », pour reprendre la terminologie si éclairante de Guy Carcassonne ; analyser l'urgence par opposition à la situation normale, celle où le respect des règles et les considérations de droit s'imposeraient parce qu'on a le temps.

Je pense notamment au report de l'installation des conseils municipaux élus au complet dès le premier tour, à la clarification des conditions de prorogation des mandats des conseillers municipaux et à l'assouplissement des modalités de réunion des assemblées délibérantes pendant la crise sanitaire. Je pense également à l'extension des prérogatives du Premier ministre pour la mise à disposition de certains médicaments et le contrôle des prix des produits nécessaires à la lutte contre l'épidémie, ainsi qu'à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire sans délai

l'état d'urgence sanitaire, l'instauration d'un régime distinct de celui issu de la loi du 3 avril 1955, inscrit dans le code de la santé publique, confère une base juridique solide et claire aux mesures prises pour lutter contre l'épidémie, assorties de sanctions et de garanties renforcées en matière de compétences, de procédures et de contrôle parlementaire. Ensuite, des mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie sont indispensables pour assurer la continuité de la vie économique et sociale éviter la défaillance des entreprises, tout en protégeant la vie, la santé et les droits des salariés. Le périmètre de ces mesures a été utilement précisé, par exemple en renvoyant à un accord collectif de branche ou d'entreprise la possibilité de réduire les délais de fixation des dates de congés payés par l'employeur, dans la limite de six jours. Je pense également aux 300 milliards d'euros de garanties d'État pour les prêts de trésorerie aux entreprises et aux 45 milliards d'euros de soutien aux entreprises, à travers notamment la suspension des principaux impôts, le report des charges sociales, le chômage partiel et un fonds de solidarité pour les TPE. Ces ordonnances, je tiens à le souligner, auront également pour objet de protéger les plus vulnérables, en particulier les personnes en situation de pauvreté, dont le dénuement et la solitude risquent d'être aggravés par la crise sanitaire.

qui doit faire l'objet d'une vigilance éclairée dans les périodes et les temporalités troublées par l'urgence, notamment à travers le contrôle du Parlement.

du Sénat tout entier, se tient aux côtés des malades et des familles touchées au coeur. Nous soutenons le personnel hospitalier, du chef de service à l'aide-soignante et au personnel chargé du nettoyage : ils sont debout, avec des moyens si faibles face à l'ampleur du mal qui s'abat. Nous saluons leur courage, leur dévouement, leur prise de risque terrible. De même, nous saluons tous les salariés, artisans et agriculteurs qui continuent à faire vivre le pays, souvent sans protection- j'y reviendrai -et sous la menace d'une remise en cause programmée de leurs droits.

n'est pas acceptable. Nous refusons de confier les pleins pouvoirs au Gouvernement pendant deux mois dans de telles conditions ! Ce qui, du reste, ne paraît pas conforme à l'esprit de la Constitution. Dans cette lutte, la démocratie est la grande oubliée- qui, dans ces moments difficiles, devrait au contraire être constamment convoquée. Notre conviction est d'autant plus forte que l'Assemblée nationale a renforcé encore les prérogatives du Premier ministre. Nous refusons refusons également l'instauration d'une sorte d'état d'urgence sanitaire de droit commun, d'une durée d'un mois, inscrit dans le code de la santé publique. Nos craintes sur les mesures sociales du projet de loi sont, elles aussi, confirmées. Nous ne sommes plus dans l'état d'urgence En effet, même si l'article 7 du projet de loi permet des accords d'entreprise ou de branche, il prévoit encore des dérogations profondes au droit du travail, qui pourront- sauf si quelqu'un me prouve le contraire maintenant ... -, s'étendre sur des années, voire devenir permanentes. Temps de travail, congés payés, travail le dimanche : dans tous les secteurs, ce sont encore une fois les salariés que vous voulez mettre à contribution pour sauver les trésoreries des entreprises, certainement pas les actionnaires ! Votre refus de rétablir l'ISF dans le projet de loi de finances rectificative est à ce titre symbolique. c'est la vie des familles, du monde du travail qu'il faut protéger. Le confinement- c'est une évidence -doit être respecté, sans écart ; mais nous désapprouvons les sanctions disproportionnées votées dans la précipitation de l'Assemblée nationale. le gouvernement italien annonce l'arrêt de toute activité de production non essentielle, Mme Pénicaud se félicite de pouvoir contraindre les salariés du BTP à reprendre le travail, tandis que M. Le Maire pousse dans le même sens en agitant l'idée d'une prime de 1 000 euros. Non !

les moyens pour l'hôpital ? Où est l'effort déterminant pour la mise à disposition de matériels ? L'inquiétude sur le manque de masques, de médicaments et de tests pour la population et même pour les personnels de santé devient criante entend-il vraiment leur désespoir ? Où sont les réquisitions d'entreprises pour la sauvegarde nationale ? Quand allez-vous rouvrir et nationaliser des sociétés indispensables, comme l'usine Luxfer, productrice du matériel pour l'oxygénothérapie ? Quand allez-vous annoncer un plan pour l'hôpital digne de ce nom ? Comme je l'ai souligné en première lecture, l'heure est à l'action et à la mobilisation générale pour la protection de tous.

ce texte, parfaitement conforme à votre projet politique, sollicite largement les travailleurs, parmi lesquels les plus exposés, alors que les forces de l'argent sont encore et toujours protégées. C'est donc en toute responsabilité que, à l'exception de deux de nos membres rattachés, nous voterons contre

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Gouvernement nous a saisis en urgence d'un projet de loi exceptionnel visant à faire face à la crise dramatique que notre pays, comme tant d'autres, traverse. Le Parlement a donc apporté sa contribution à la lutte contre le virus, comme tous les Français apportent la leur. Je tiens d'abord, comme nos concitoyens le font désormais tous les soirs à

La situation est grave, mais nous la surmonterons, à une condition : rester unis et solidaires. Car, comme on nous l'a appris il y a des siècles, toute demeure divisée périra. Il nous fallait d'abord nous donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Personne n'aurait compris que nous n'y arrivions pas ensemble. Avec nos collègues députés, nous sommes donc parvenus à un texte commun. Il fallait nous donner des moyens, mais aussi garantir le respect du droit. Ce texte consacre la création d'un régime d'état d'urgence sanitaire, prévoyant notamment la possibilité de réquisitionner toutes les personnes et tous les matériels nécessaires à la lutte contre le virus. permet aussi d'encadrer, pour des raisons sanitaires, l'ouverture des commerces et les déplacements de nos concitoyens. Ces mesures sont radicales, mais c'est la condition de leur efficacité. Dans une démocratie comme la nôtre, toutefois, il est essentiel de veiller à leur contrôle. C'est donc le Parlement qui décidera de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Les fermetures de lieux de vie et de commerces et les mesures de confinement, qui impliquent un contrôle accru de nos frontières, ont pour objectif de ralentir la propagation du virus et d'éviter la saturation des hôpitaux. Mais ces mesures ont aussi des effets redoutables sur l'économie. Les médecins savent qu'il y a des remèdes pires que le mal. De là leur devise, : avant tout, ne pas nuire. C'est la raison des mesures exceptionnelles que nous devons prendre pour soutenir l'économie.

ralentir les autres activités pour limiter sa propagation. Il faudra donc suspendre largement les délais, ceux qui pèsent sur les entreprises, bien sûr, mais aussi tous les autres : forclusion, prescription, déchéance et nullité. cette suspension ne doit pas signifier la paralysie de notre pays. Il faut continuer de travailler, de produire. Il faut aussi assurer la continuité de nos services. Les allocations ou les prises en charge dues à nos concitoyens doivent continuer d'être versées malgré la crise- ou plutôt, à cause de la crise. L'épidémie de coronavirus a fortement perturbé la tenue des élections municipales. Le projet de loi comporte les adaptations nécessaires au bon fonctionnement des institutions locales. L'épidémie que nous traversons est une épreuve redoutable, mais, comme le disent les Anglais, une mer calme n'a jamais fait un bon marin ... Grâce à notre détermination et à notre créativité, nous pouvons faire de cette crise une opportunité de nous dépasser et de nous renforcer. Ce projet de loi marque une avancée importante dans la résolution de la crise. Le groupe Les Indépendants le soutient pleinement. « Le commencement est la moitié du tout », disait Aristote. Nous avons commencé. Et nous nous tenons prêts, dès aujourd'hui, avec l'ensemble de nos collègues, à accompagner le Gouvernement dans la suite de ce combat Nous avons tous conscience des contraintes que créent les décisions que nous prenons aujourd'hui. Nous allons imposer aux Français l'obligation de la patience. Chacune et chacun d'entre eux va devenir pour quelques semaines un Robinson Crusoé. Les rivages de notre île seront les murs de nos maisons ou de nos appartements. Certains y vivront seuls, d'autres auront la chance de les partager avec un ou plusieurs Vendredi. À mesure que les jours succéderont aux jours, une forme de routine étrange va s'installer pour les Français. Ce sera dur pour eux, car ils sont plus obstinément attachés à leur liberté qu'ils ne sont naturellement doués de patience. Ils vont devoir s'adapter à une situation contre nature, contre leur nature, et faire confiance à leur allié dans ce combat : le temps. Jusqu'à ce jour, le temps était un ennemi, du moins un adversaire. Notre époque, qui est plutôt celle de la fulgurance, confond volontiers le rapide et le vivant. Nous vivons au temps du haut débit et du train à grande vitesse. Nous avons même appris à multiplier le temps, ou plutôt les tâches nous travaillons sur nos ordinateurs tout en dialoguant par WhatsApp avec des amis et en consultant nos mails, le tout sur fond d'un concerto de Mozart. Le problème, avec la recherche de l'intense, c'est qu'elle ruine la sensibilité et l'intimité. Nous ne recherchons plus le calme, parce qu'il nous semble un sommeil ... Je voudrais proposer aux Français de profiter de ces quelques semaines d'isolement forcé pour partir, comme nous le suggérait Proust, à la recherche du temps perdu. Tout le monde connaît la première phrase de son oeuvre : « Longtemps, je me suis couché de bonne heure. » Nous allons pouvoir nous coucher et nous lever à l'heure que nous voulons et retrouver pendant un moment la maîtrise de nos journées. Nous allons pouvoir penser, car, comme le dit le Bouddha, « la patience est la plus grande des prières ». Peut-être même parviendrons-nous à mettre en pratique cet aphorisme de Vauvenargues : « La patience est l'art d'espérer. » Car, en définitive, la seule chose dont les Français aient besoin en ce moment, c'est l'espoir.

les médecins, qu'ils soient expérimentés ou jeunes internes. Tous sont mobilisés pour faire face à un défi sanitaire sans précédent dans notre pays. J'ai une pensée toute particulière pour ce médecin dont on a appris le décès aujourd'hui dans l'Oise.

Le Président de la République s'est exprimé à deux reprises en moins d'une semaine. Son message était sans équivoque : nous sommes en guerre ; en guerre contre une menace invisible, mortifère, sournoise, un virus qui touche tout le monde et prend des dimensions graves ou dramatiques chez les personnes les plus âgées et les plus vulnérables, un virus qui met au défi l'ensemble de notre système de santé, l'un des plus performants au monde, un virus qui, depuis lundi soir, a bouleversé radicalement, et pour longtemps, le quotidien de tous nos compatriotes, un virus qui met aussi en péril toute notre économie, nos entreprises, leurs salariés, nos artisans, nos commerçants, nos travailleurs indépendants et nos agriculteurs. Je veux saluer à mon tour ces millions de Français qui, malgré les circonstances, continuent à aller travailler, parce que leur activité est indispensable à la vie du pays dans les services publics, l'agroalimentaire, la grande distribution, les transports, l'énergie ou encore la gestion des déchets. Il faut les remercier, mais aussi s'assurer qu'ils ne mettent pas leur propre vie en danger en leur apportant toutes les protections nécessaires. Il est important- et je crois, monsieur le président, que vous avez saisi le Premier ministre ou le Président de la République -que le Gouvernement clarifie sa démarche. D'un côté, on demande à nos compatriotes de demeurer en confinement. Ils ont commencé à entendre ce message, et la plupart d'entre eux le respectent ; de l'autre, on demande à certains d'aller travailler.

Nous saluons la décision du Gouvernement de supprimer le jour de carence. Nous avions très tôt insisté sur ce point, et nous sommes rassurés d'avoir été entendus. Il nous faut dès à présent anticiper la sortie de crise, car sortie de crise il y aura, évidemment. Après le séisme sanitaire, nous ne pouvons pas nous permettre un tsunami économique, qui mettrait durablement des millions de Français au chômage, qui installerait la précarité et la paupérisation de pans entiers de notre société avec, au milieu, un État financièrement exsangue. La relance, la reprise doivent se préparer dès maintenant. Elles doivent être coordonnées, bien sûr au niveau européen, mais aussi mondial. Nous souhaitons ainsi que le Gouvernement informe régulièrement le Parlement sur la stratégie qu'il entend mettre en oeuvre après la levée du confinement, ce confinement dont certains de nos concitoyens ne semblent pas toujours avoir compris l'importance cruciale. Inconscients de l'ampleur de la menace que constitue cette épidémie, ils ne veulent pas tenir compte des consignes. Pour ceux-là, qui mettent en danger leur vie, mais surtout celle des autres, la réponse de l'État doit être ferme, très ferme. Le texte que nous votons permettra de sanctionner ces comportements irresponsables. Ce virus a également bouleversé nos institutions et le fonctionnement de notre démocratie. Nous devrons en tenir compte, monsieur le président : il faudra que nos assemblées réfléchissent aux moyens de poursuivre leurs activités lorsque nous avons à faire face à un fléau comme celui d'une épidémie. On a vu combien nous étions démunis et devions, jour après jour, sous votre autorité, adapter notre mode de fonctionnement.

Je me félicite de l'état d'esprit républicain qui a animé l'ensemble de nos collègues, sur quelque travée qu'ils siègent, et je veux vous remercier, monsieur le président, de la concertation de qualité que vous avez su organiser avec l'ensemble de nos groupes. Nous avons pleinement exercé notre rôle de législateur- cela était indispensable -, tout en apportant un soutien sans équivoque aux actions lancées par l'exécutif. À mon tour, je signale que notre groupe, bien évidemment, soutiendra par son vote le texte. Il me reste à saluer le président Bas pour la qualité du travail qu'il a réalisé dans des circonstances particulièrement difficiles

voici plus d'une semaine que la France vit à un rythme ralenti. L'épidémie de Covid-19 est devenue la plus grande crise de santé publique dans notre pays depuis un siècle. Pour faire face à ces circonstances difficiles, le Parlement a été saisi dans l'urgence d'un projet de loi organique et d'un Compte tenu de la gravité de la situation, le Sénat a travaillé en lien très étroit avec le Gouvernement et l'Assemblée nationale. Nous avons préparé en quatre jours une loi qui offrira aux autorités publiques et à la société tout entière des outils puissants et flexibles dans leur riposte face au virus.

Cet impératif a fait l'objet d'un large consensus parmi toutes les forces politiques. Le Sénat l'a fait sien, et la commission mixte paritaire l'a confirmé, en aboutissant à un texte de compromis. Que contient le texte final du projet de loi ? D'abord, il crée l'état d'urgence sanitaire. Cet état donne au Gouvernement la possibilité de prendre par décret des mesures exceptionnelles, couvrant des domaines énumérés par la loi. restreindre la liberté d'aller et venir, ordonner la mise en quarantaine, la fermeture provisoire de certains établissements, ou encore limiter les rassemblements sur la voie publique. Il s'agit là de mesures hautement dérogatoires au droit commun, mais justifiées au regard des circonstances. La loi comprendra aussi des garanties de proportionnalité et de contrôle par la justice et le Parlement. Cela doit permettre d'assurer l'équilibre entre les droits et libertés, d'une part, et les nécessités s'imposant à une société menacée par l'épidémie, d'autre part. Ces derniers jours, certains individus ont pu, sciemment, se défier des obligations de confinement, mettant ainsi en danger, par inconscience ou par égoïsme, la grande majorité de nos concitoyens, qui, par civisme et respect de leur prochain, respectent les préconisations sanitaires. Cet état d'urgence permettra aux forces de l'ordre, y compris les polices municipales, de mieux sanctionner de telles actions, qui plus est, avec une sévérité accrue en cas de récidive. Enfin, le Sénat a veillé à garantir que ce dispositif ne perturbe pas l'équilibre des pouvoirs, et cela en se prononçant pour un contrôle parlementaire attentif de l'ensemble des mesures prises par le Gouvernement sous cet état d'urgence sanitaire. Il s'est aussi assuré que ce dernier demeure strictement temporaire et ne devienne pas un nouveau régime d'exception durablement inscrit dans notre droit. Ensuite, la nouvelle loi habilitera le Gouvernement à prendre un grand nombre d'ordonnances afin d'adapter la vie économique, sociale et administrative à une France largement confinée. Vous connaissez tous, chers collègues, notre réticence face au recours trop large aux ordonnances. Dans un monde idéal, nous disposerions du temps nécessaire pour discuter de chaque mesure à prendre, peser le pour et le contre et voter un texte. Malheureusement, ce n'est pas là une approche réaliste quand des Français décèdent chaque jour de ce virus. Pour cette raison, il est raisonnable d'habiliter le Gouvernement à agir tout de suite et rendre vite possible l'adoption des mesures provisoires qui s'imposent. Les entreprises, les salariés, les indépendants, les administrés ont besoin d'aide et d'options dès maintenant. Enfin, la loi Urgence Covid permettra de résoudre l'essentiel des difficultés concrètes auxquelles font face les collectivités, qui sont prises dans une sorte de purgatoire entre les deux tours des élections municipales. Cet état, parfaitement anormal au regard de notre droit, risquerait, s'il se poursuivait, de désorganiser la capacité de nos élus locaux et de leurs équipes à faire face à l'épidémie sur le terrain. Sans entrer dans le détail des différentes mesures, la loi offrira de la clarté sur le destin des conseils municipaux déjà élus. Ceux-ci pourront entrer en fonction une fois que le Gouvernement, informé par le conseil scientifique, estimera que les conditions sanitaires rendent la première réunion possible. D'autres dispositions permettront aux collectivités de fonctionner politiquement, administrativement et financièrement jusqu'au deuxième tour. Pour conclure, je tiens à saluer une nouvelle fois le courage, l'abnégation et le sens du sacrifice de tous ceux qui participent à la défense de la société française contre la maladie : les personnels soignants et de sécurité, évidemment, mais aussi les nombreux travailleurs des secteurs critiques où le confinement n'est pas possible- caissières, routiers, personnels techniques de l'énergie, des transports, et bien d'autres. Le projet de loi que nous allons voter aujourd'hui doit être un moyen de leur dire vous qui êtes au front, soyez assurés que nous sommes tous derrière vous et que nous n'avons reculé devant rien pour vous apporter toute l'assistance dont vous avez besoin. L'heure n'est pas aux atermoiements, elle est à l'action ! Le Parlement a joué son rôle et a donné au Gouvernement des moyens extraordinaires pour faire face à la crise. À présent, c'est à ce dernier de se montrer à la hauteur. Vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains votera ce texte et surveillera attentivement tant la mise en oeuvre de l'état d'urgence que le contenu des ordonnances à venir.

un peu comme en temps de guerre- même si les circonstances sont différentes -, notre liberté de mouvement, notre liberté d'action ne sont pas celles dont nous disposons en temps ordinaire. Pourtant, il est essentiel de les préserver. En légiférant,

sur tous les aspects de ce texte. Or ne reste plus dans la version que nous allons adopter qu'une information particulière sur l'état d'urgence sanitaire, mais pas sur les mesures économiques et sociales. Par ailleurs, ce projet de loi comporte le renvoi à de nombreuses ordonnances. Pour ces deux raisons,

commissions concernées : le président de la commission des affaires sociales, la présidente de la commission des affaires économiques et moi-même. Si vous avez la bénévolence d'accepter de prendre cet engagement, je suis persuadé que le président de notre assemblée

associés au travail qui s'effectuera sur la base des informations que vous nous donnerez.

monsieur le président, mais n'agissons pas à la légère. Il ne s'agit pas de mesures anodines : elles limitent la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion, la liberté d'entreprendre. Elles concernent le fonctionnement même de la démocratie représentative. Elles mettent en cause certains principes et acquis de notre droit du travail. ce sujet, de remercier à mon tour les millions de Françaises et de Français qui font vivre notre pays en cette période. Une crise, quelle qu'elle soit, ne peut servir de prétexte à affaiblir durablement les principes démocratiques fondamentaux, les libertés publiques et individuelles, le socle social de notre démocratie. Un état d'exception est par définition attentatoire aux libertés- tel est l'objet même d'un état d'exception. Mais, sous peine de renoncer à notre identité, il faut répliquer avec les moyens attachés à l'État de droit, dont fait partie, monsieur le président, le contrôle du Parlement, que nous voulions plus fort, notamment dans l'association à l'élaboration des ordonnances. J'ai bien entendu votre message, monsieur le ministre. Il se trouve que nous avons un peu de temps pour vous aider dans l'élaboration des ordonnances en cette période La Constitution est notre ultime refuge. Elle sait s'adapter aux jours de tempête comme aux jours de miel, pour reprendre la belle expression d'Albert Camus. Comme la démocratie, elle est une arme dans cette crise. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste et républicain demande en premier lieu au Président de la République de saisir le Conseil constitutionnel de cet objet non identifié, qui ne peut, qui ne doit ressembler ni de près ni de loin à un article 16 rampant à caractère sanitaire. J'espère aussi qu'à l'occasion de cette crise le Gouvernement comprend que nos agents publics et nos services publics sont nécessaires au fonctionnement du pays. Ils doivent être considérés comme une chance et non comme un coût. Il est temps de mettre un terme à la gestion d'apothicaire qui constitue votre politique en la matière. Cette crise doit également conduire à une refonte de la politique industrielle. Je pense en particulier à la réimplantation d'entreprises à caractère stratégique, notamment en matière de médicaments. Cette crise, je l'espère, sera enfin l'occasion de renouer avec les corps intermédiaires à l'issue d'une période autoritaire. La qualité du dialogue social sera l'une des conditions de reconstruction du pays, la condition d'une confiance retrouvée. N'ayons pas peur de la démocratie sociale. Nous y prendrons toute notre part. Nous sommes favorables au principe de l'état d'urgence sanitaire, même si nous regrettons que le Gouvernement n'ait pas pris en compte nos remarques qui visaient à garantir l'unité nationale face à l'épidémie. Viendra ensuite l'heure du bilan. D'ici là, en responsabilité, nous vous confirmons que nous allons nous abstenir sur ce projet de loi.

-, Jacques Oudin a été élu en Vendée, sur la petite île de Noirmoutier. Il a été un grand parlementaire, un grand sénateur de la République française.

Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous voterons ce texte, parce que nous ne voulons pas entraver l'action du Gouvernement et parce qu'il nous semble que cet état d'urgence sanitaire doit être mis en oeuvre le plus vite possible.

-prévoyant que les autorités administratives communiquent toute mesure prise ou mise en oeuvre en application de la loi à l'Assemblée nationale et au Sénat et que le Parlement peut requérir toute information complémentaire en ce qui concerne le contrôle et l'évaluation de ces mesures ainsi que les conséquences sanitaires

orateurs ont estimé que ce dernier était disproportionné par rapport à la situation actuelle. Pourtant, l'article 16 prévoit d'associer étroitement le Parlement et le Conseil constitutionnel à la mise en oeuvre Vous avez choisi de créer un nouveau régime d'exception, qui n'offre pas les mêmes garanties de consultation et de préservation des droits du Parlement et des libertés individuelles. Ce choix discutable doit être discuté, notamment par le Conseil constitutionnel. À tout le moins, il vous oblige à associer encore plus étroitement à la gestion de cette crise le Parlement et les juridictions administratives. Face à l'épidémie, la République doit s'unir, certes, mais pas sous la seule autorité de l'exécutif. Toutes les composantes de la Nation doivent être associées dans un effort collectif et citoyen. Notre groupe veillera avec détermination au respect strict des principes constitutifs de la République. La

face à l'urgence sanitaire, sociale et humaine. Au terme de ces quatre jours, nous sortons de cette session avec un goût amer, parce que le travail effectué n'est pas à la hauteur de la situation. Souvenez-vous que nous avons adopté un projet de loi de finances rectificative, qui débloque des sommes importantes pour aider l'économie- objectif que nous partageons

les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre I de la troisième partie du code du travail,

Nous connaissons trop bien la tentation qui consiste à faire payer ce type de crise aux petits, et nous n'accepterons pas qu'il en soit ainsi

certes rapide, mais efficace. Nous restons, nous l'avons dit, insatisfaits des moyens qui seront donnés au Parlement, notamment au Sénat, pour contrôler l'action du Gouvernement. Pour autant, nous sommes disponibles et tout à fait mobilisés

puissent continuer à fonctionner et que le Sénat et l'Assemblée nationale assument pleinement leurs missions, dont la continuité est indispensable au bon fonctionnement de notre démocratie parlementaire.

comme je vous l'avais indiqué lors de notre précédente séance publique, nous maintiendrons, ainsi que l'a décidé la conférence des présidents, des séances de questions au Gouvernement le mercredi à quinze heures dans un format restreint